Madame la ministre, mes chers collègues, il nous reste 141 amendements à examiner sur ce texte. Je vous propose d'ouvrir la soirée, qui était éventuelle, et la nuit, pour achever l'examen des articles. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé.

qualifiées par l'auteur du de « tyrannie à mille têtes [ ...], meilleure forme que l'oppression ait jamais pu prendre pour écraser les individus et les intérêts généraux ». Ne

dotés d'autorités organisatrices, que ce soit l'État ou les régions. Nous ne croyons pas en un système où se côtoient un service régulé et un service strictement concurrentiel. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

l'avis du Gouvernement ? Madame Assassi, j'ai bien compris que vous étiez opposée à l'ouverture à la concurrence. Mais, en l'occurrence, l'article 2 réaffirme le rôle de l'État comme autorité organisatrice compétente pour l'organisation des services de transport ferroviaire d'intérêt national, national, la possibilité de conclure des contrats de service public pour exploiter des services d'intérêt national et le rôle des régions comme autorités organisatrices des services régionaux.

de l'alinéa 3 de l'article 2 , « les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national et les services de transport routier effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires » sont assurés par les entreprises ayant conclu avec l'État, autorité organisatrice, un contrat de service public. Peu importe le type de contrat conclu entre l'État et l'autorité organisatrice des services de transport routier : nous sommes opposés à ce que les services de transport ferroviaire d'intérêt national puissent être assurés durablement par des autocars.

Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour l'État de conventionner des services routiers effectués en substitution de services ferroviaires. Certes, je comprends et partage les réserves des auteurs de l'amendement sur le report des services ferroviaires sur la route, mais il y a des cas où le recours au transport routier est plus pertinent,

Il s'agit d'articuler au mieux les services conventionnés et les services librement organisés. Il est prévu de permettre aux régions de conventionner des services au-delà de leurs frontières, mais il faut veiller à ce que ces services ne remettent pas en cause l'équilibre économique de services librement organisés, car les modèles économiques des opérateurs peuvent être fragiles. C'est une règle de protection symétrique de celle pour les services conventionnés, à cette différence notable près que l'avis qui pourra être demandé à l'ARAFER ne sera qu'indicatif. Cet avis aura l'intérêt d'éclairer la région sur les conséquences de son projet, par exemple dans le cas où une offre conventionnée supplémentaire

? Cet amendement vise à rétablir une disposition que nous avons supprimée en commission : l'interdiction faite aux régions de conventionner des services au-delà de leur ressort territorial s'ils portent atteinte à l'équilibre économique des services commerciaux. Il faut tout d'abord relever que la logique d'une telle disposition est complètement inverse de celle du droit européen. Celui-ci vise au contraire à préserver l'équilibre économique des services conventionnés par rapport aux services commerciaux dans le cadre du libre accès au réseau. outre, la mesure semble inutile. Dans le contexte financier actuel, les régions n'auront pas d'intérêt à subventionner des services effectuant des liaisons identiques à celles qui sont assurées par des services commerciaux qui sont rentables sans subvention. Cela va de soi telle disposition pourrait limiter les possibilités des régions de conclure des contrats de service public incluant des services rentables et des services non rentables. Or cela n'est pas souhaitable, dans la mesure où ce mécanisme permet de garantir des dessertes directes sans correspondance, ce à quoi nous sommes très attachés. La

Monsieur le rapporteur,

Il s'agit parfois d'un accord global sur le schéma de desserte TGV d'un territoire. Il peut également s'agir d'autoriser les abonnés des TER à emprunter certains TGV pour des dessertes au sein de la région. Une desserte TGV bien articulée avec l'offre TER permet de proposer aux abonnés régionaux un service rapide et confortable entre les grands pôles d'une même région. Pour ce type de desserte, il peut y avoir complémentarité entre les offres TER et TGV. Une telle organisation de l'offre de services a un double avantage : d'une part, la région peut programmer moins de TER en utilisant les capacités disponibles des TGV ; d'autre part, la SNCF peut s'assurer un meilleur remplissage de ses TGV.

Ces deux amendements identiques sont très intéressants. Ils concernent les contrats de service public conclus avec des entreprises offrant un service de voyageurs librement organisé pour qu'elles adaptent les conditions d'exploitation du service ou qu'elles autorisent la montée à bord de voyageurs régionaux.

Je voudrais rappeler à ce sujet que le droit européen n'autorise la conclusion de ces contrats qu'après une procédure de mise en concurrence dans les règles. Cela est précisé dans les deux amendements. Dans ce contexte, je ne suis pas opposé à ce que l'ARAFER vérifie si les compensations demandées ne sont pas excessives compte tenu de la faible concurrence attendue, dans un premier temps, pour les services librement organisés. La commission émet donc un avis

est à Mme la ministre. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu : je partage tout à fait la préoccupation de mieux coordonner les offres de transport.

L'ARAFER estime, dans sa contribution de mars 2018, que « l'évaluation correcte du niveau actuel de rentabilité des services commerciaux est impossible en l'absence d'une séparation comptable des activités de SNCF Mobilités ». par SNCF Mobilités, une comptabilité analytique par liaison des services non conventionnés, afin d'obtenir une base chiffrée pour l'établissement des politiques publiques de transport. L'amendement vise à imposer à SNCF Mobilités d'établir une comptabilité analytique par liaison de l'ensemble des services non conventionnés d'ici au 1 janvier 2020. Il apparaît paradoxal de lui imposer une telle norme pour les services commerciaux qui ne font pas l'objet de financements publics, au moment même où elle va se trouver en concurrence avec les autres entreprises ferroviaires, qui ne seront pas soumises à la même règle.

Nous craignons en effet que, faute de volonté politique, ces lignes ne fassent pas l'objet de contrats de service public. L'État ne les conventionnera pas, laissant ainsi aux régions le choix de les reprendre ou non. Les régions n'auront alors d'autre option que de reprendre ces lignes ou de les supprimer. Certaines lignes de TER risquent également de faire les frais de ces nouveaux contrats de service public. En réalité, vous allez étouffer un tiers du réseau en faisant assumer cette responsabilité par les régions, qui auront mission de trouver des opérateurs acceptant d'assurer la circulation sur ces petites lignes. Autant dire qu'elles n'y parviendront pas, ou difficilement, et qu'elles ne lanceront leurs appels d'offres qu'après avoir assaini- c'est-à-dire atrophié -le réseau, pour ne maintenir que les lignes rentables. On nous expliquera ensuite que les régions ne pouvaient pas tout financer- ce qui n'est pas faux -et qu'il était nécessaire de faire des choix pour maintenir un service de qualité sur les tronçons les plus fréquentés. Cet article ouvre donc la voie à une diminution du service public ferroviaire, quelles que soient

Alors même que ces trains transportent quotidiennement toutes les catégories de populations, les personnes qui étudient, celles qui travaillent, celles qui vont se faire soigner, celles qui voyagent, serons-nous amenés à leur dire un jour : désolés, il n'y a plus de train ? des transports du quotidien, qui doivent être rénovés et modernisés, l'exécutif, qui en fait supporter toute la charge aux régions Il y va de la façon dont nous voulons aménager notre territoire et assurer la qualité de son maillage. Par exemple, on a beaucoup parlé de la ligne Abbeville-Le Tréport, qui va être fermée faute d'accord entre l'État, la région Normandie et ma région, les Hauts-de-France. Pour la petite histoire, la gare d'Abbeville, construite en 1855, vient d'être

l'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer : soit lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau concernés et notamment leur taille, les caractéristiques de la demande, la complexité du réseau, son isolement technique et géographique et les services couverts par le contrat soit lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux, par rapport au précédent contrat ». La CGT indique, dans son document, qu'en s'appuyant sur son document, qu'en s'appuyant sur ce texte et en exigeant des normes sociales, qualitatives et environnementales de haut niveau, comme prévu au paragraphe 6 de l'article 4, la Nation peut garder le service public ferroviaire. Nous partageons largement cette analyse

l'initiative du rapporteur, la commission a adopté une nouvelle rédaction de l'article 4 , relatif à la transmission des données couvertes par le secret professionnel et commercial. Ainsi, le rapporteur a étendu l'obligation de transmission à l'ensemble des informations relatives « à l'organisation ou à l'exécution de ces services et aux missions faisant l'objet du contrat de service public, et non aux seules données nécessaires à la préparation d'une procédure de mise en concurrence

L'ouverture à la concurrence ne doit pas permettre aux nouveaux entrants de récupérer des savoir-faire et des informations confidentielles sans aucune réciprocité, leur conférant d'entrée de jeu un avantage concurrentiel sur l'opérateur historique. Dans de telles conditions, l'ouverture à la concurrence peut affaiblir et remettre en cause, à terme, la viabilité de ce dernier. Loin d'être libre et non faussée, la concurrence risque d'être déloyale si elle est bâtie sur une asymétrie d'information à l'avantage des nouveaux entrants.

apporter un certain nombre de précisions sur les conditions de transmission des données. Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 traite

que l'opérateur choisi doit fournir tout au long de l'exécution du contrat. Les premières relèvent de la loi et de l'obligation qui est faite à l'opérateur sortant, les secondes

un équilibre. Les auteurs de l'amendement n° 200 souhaitent revenir sur le principe de la transmission aux autorités organisatrices d'informations couvertes par le secret industriel et commercial. Le souci de protéger ces informations est tout à fait légitime, mais il faut aussi avoir à l'esprit que la transmission de certaines données couvertes par le secret est indispensable pour que l'autorité organisatrice puisse définir correctement le périmètre de son appel d'offres, apprécier l'équilibre économique du contrat et garantir le caractère équitable et non discriminatoire de la procédure de mise en concurrence. L'ARAFER a d'ailleurs clairement affirmé cette nécessité. Je relève que le projet de loi initial prévoyait déjà la transmission de données couvertes par le secret industriel et commercial. La rédaction adoptée par la commission a établi un équilibre entre ces deux préoccupations légitimes : elle a certes élargi le champ des données à transmettre aux autorités organisatrices, mais elle a aussi, en parallèle, renforcé la protection des informations couvertes par le secret industriel, en prévoyant l'application de l'article 226-13 du code pénal en cas de divulgation de ces données à des tiers non autorisés. Par ailleurs, la communication de certaines de ces informations aux candidats à un appel d'offres est aussi nécessaire pour éviter que l'opérateur historique ne bénéficie d'une rente informationnelle lui donnant un avantage concurrentiel par rapport aux nouveaux entrants. Je rappelle que le dispositif adopté par la commission est proportionné et encadré cette communication n'aura lieu que lorsqu'elle est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'ARAFER, pour protéger la confidentialité de ces données. avons prévu ceinture et bretelles ! Certaines informations devront, par exemple, être présentées par fourchette de valeurs ou ne pourront être consultées que dans une salle spécifique.

de l'exécution des contrats pour en assurer le suivi. Je m'appuie, là encore, sur la contribution de l'ARAFER sur l'ouverture à la concurrence des services conventionnés. Nous connaissons trop

mentionne la possibilité de transmettre ces informations, mais de façon très encadrée, me semble constituer un bon équilibre. Par conséquent le Gouvernement

une précision qui n'aurait qu'une valeur indicative, permettant à l'autorité organisatrice de détecter, en amont, les sujets sur lesquels il pourrait y avoir divergence, donc contentieux, en cas de transmission.

Nous contestons ce pouvoir d'autorisation confié à l'ARAFER. En effet, nous le savons tous, le rôle et la raison d'être de cette autorité indépendante sont de faire de la place aux nouveaux entrants. C'est d'ailleurs cette même autorité qui avait déclaré que, si prise isolément, chacune des dérogations autorisées par le quatrième paquet ferroviaire peut présenter un intérêt opérationnel, leur application cumulée pourrait faire peser un risque de ralentissement du processus d'ouverture à la concurrence, à rebours de l'esprit de ce quatrième paquet ferroviaire.

que, lorsque la procédure est d'attribution directe, conformément aux paragraphes 3 4, 4 et 4de l'article 5 du règlement OSP, le contrat de service public doit être attribué à l'opérateur historique. Aujourd'hui, SNCF Mobilités est en situation de monopole. Demain, il u aura des opérateurs concurrents. Permettre, dès la phase d'ouverture à la concurrence, d'attribuer directement un contrat de service public, c'est-à-dire sans recourir à une procédure de mise en concurrence,

pour encadrer le recours à certaines exceptions à l'obligation de mise en concurrence prévues dans le règlement OSP. La disposition qui a été adoptée en commission va au-delà de l'obligation d'évaluation par un organisme indépendant prévue par les textes. Les garanties de transparence, avec une évaluation préalable de l'ARAFER et la possibilité d'en appeler au juge avant l'attribution directe, me semblent suffisamment dissuasives pour prévenir tout comportement

et à recourir, dans les cas prévus par l'article 5 du règlement européen OSP, à la procédure d'attribution directe. Il conditionne cependant le choix de l'AOT d'utiliser ces dérogations à l'avis de l'ARAFER lorsque celle-ci est saisie par

Le règlement OSP prévoit un certain nombre de dérogations à l'obligation de mise en concurrence des services conventionnés, que les États membres sont libres d'autoriser ou non dans leur droit national. Certaines de ces dérogations sont bien délimitées et ne posent pas de problème. C'est le cas de celle qui est prévue pour les contrats de moins de 7,5 millions d'euros ou de moins de 500 000 kilomètres de service.

161. L'amendement n° 250 vise à préciser que lorsqu'une autorité organisatrice attribuera directement un contrat après 2023, en application des dérogations prévues par le règlement européen, elle l'attribuera à SNCF Mobilités.

L'amendement n° 199 tend à supprimer la possibilité, pour toute personne à qui la décision fait grief, de saisir l'ARAFER pour évaluer le recours à la dérogation à l'obligation de mise en concurrence prévue au 4 de l'article 5 du règlement européen. Cette dérogation concerne des portions très limitées du réseau ferré national sur lesquelles les services peuvent être assurés par un opérateur qui gère aussi l'infrastructure. Les auteurs de l'amendement évoquent une surtransposition du droit européen, mais le règlement européen prévoit bien, au 7 de son article 5, « la possibilité de demander que la décision motivée prise par l'autorité compétente fasse l'objet d'une évaluation par un organisme indépendant désigné par l'État membre concerné », notamment pour la dérogation prévue à l'article 4. C'est exactement ce que prévoit l'alinéa 11. La commission ne souhaitant pas revenir sur cette disposition qui est conforme au droit européen, l'avis est défavorable.

le redis, il s'agit d'une dérogation qui concerne des portions très limitées du réseau ferré national, sur lesquelles les services peuvent être assurés par un opérateur qui gère aussi l'infrastructure. Il s'agit, d'après les services du ministère, des lignes à voie métrique Saint-Gervais-Vallorcine, dans la vallée de l'Arve, dite du « train jaune », en Occitanie,

Il me semblait aller de soi que l'évaluation faite par l'ARAFER avait un caractère consultatif, puisque, pour les deux autres dérogations, prévues au 3 et 4 , nous avons prévu un avis conforme. Cependant, je ne suis pas opposé à une telle précision.

détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.

Je pense que nous devons avoir un débat argument contre argument, extrêmement politique. Nous abordons ici la question du « sac à dos social », qui est censé permettre aux cheminots de continuer à bénéficier de leurs droits, même en cas de changement d'opérateur si la SNCF perd les appels d'offre pour les lignes ouvertes à la concurrence. Là encore, cet article, inséré par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, n'a fait l'objet ni d'une étude d'impact ni d'un avis du Conseil d'État. Nous le regrettons profondément.

Premièrement, les règles instaurées ne s'appliqueront que pour les salariés dont l'expérience dans l'entreprise est supérieure à six mois. On peut en déduire que, pour les autres, ce pourra être le licenciement en cas de perte du contrat de service public. Deuxièmement, les conséquences du refus d'un agent de la SNCF de changer d'employeur ont été précisées en commission. Pour autant, ce refus pourra, dans certains cas, constituer un motif de fin de contrat. de fin de contrat. Nous ne pourrons jamais accepter cela ! Certes, le volontariat est privilégié, mais il faut également permettre aux cheminots qui le souhaitent de conserver leur emploi au sein de la SNCF ou, pour le moins, créer une réelle obligation de reclassement pour l'entreprise historique. Les agents de la SNCF ne souhaitent pas forcément travailler au sein d'une entreprise privée, car ils sont attachés à l'opérateur historique. Si cette possibilité n'est pas expressément prévue, la prétendue « garantie de l'emploi » ne sera qu'un mensonge supplémentaire. Pour cette raison, nous demandons également un réel droit au retour au statut pour les cheminots. Par ailleurs, grâce à ces processus de transfert, les opérateurs privés vont disposer de salariés dont le coût de la formation aura été assumé par l'opérateur public. C'est un avantage non négligeable. Que dire également de la situation au sein des opérateurs privés, qui compteront en définitive deux catégories de salariés : ceux qui bénéficient du maintien de leurs garanties sociales et les autres, ceux qui n'auront pas eu la chance d'être passés par la SNCF Plusieurs questions restent en suspens. Que se passera-t-il si la ligne sur laquelle le cheminot travaille est abandonnée à l'échéance du contrat de service public par la région ? Jusqu'à quelle échéance pouvez-vous réellement garantir la poursuite de la mise en oeuvre de ce sac à dos social ? Il y a trop d'ambiguïté et de silence coupable. Cela nous conduit à nous opposer à cet article. Je veux remercier

En effet, cet article, inséré à l'Assemblée nationale, définit les règles de transfert des personnels de la SNCF en cas de reprise de l'exploitation du réseau ferroviaire par des opérateurs privés. Nous contestons tout autant la méthode que le fond. Ainsi, la méthode utilisée par le Gouvernement est particulièrement discutable. vous sortez ce projet de loi d'habilitation pour ensuite négocier avec les partenaires sociaux. C'est l'inverse qu'il aurait fallu faire : prendre le temps de négocier, pour ensuite présenter un projet de loi en bonne et due forme au Parlement. Nous nous trouvons placés dans une course contre la montre, ce qui ne crée pas les conditions d'un travail parlementaire de qualité. D'ailleurs, on voit bien que tout n'est pas ficelé, puisque des négociations ont encore lieu, comme en témoigne le nombre d'amendements présentés par le rapporteur par le rapporteur en commission, amendements qui sont plus acceptables que les dispositions initiales. Certains points nous semblent particulièrement inacceptables. Si le projet de loi fonde les transferts sur le volontariat, la problématique du refus du salarié reste posée. Nous considérons, pour notre part, que le refus est un droit du salarié et que son expression ne doit pas avoir d'incidence sur la poursuite du contrat de travail. Trop d'incertitudes demeurent encore sur les conditions de reprise, sur les garanties sociales. Enfin, quelle aubaine, disons-le, pour les entreprises privées de pouvoir embaucher un personnel qualifié et compétent sans avoir eu à supporter le coût de sa formation. Encore un cadeau qui est fait aux nouveaux entrants ! Ils récupèrent le matériel roulant, les ateliers de maintenance et les personnels ! C'est tout de même incroyable ! Voilà une belle opération Nous entendons que toutes les garanties soient données aux cheminots. Dans l'attente d'un dialogue social fructueux, et prenant acte que, dans leur très grande majorité, les cheminots sont opposés à la présente réforme, nous demandons la suppression de cet article.

que les droits garantis aux salariés transférés. Le transfert de personnel, lorsqu'une entreprise succède à une autre entreprise, est un principe appliqué dans de nombreux secteurs d'activité, par exemple dans celui des transports urbains. Cette obligation de reprise des salariés par le nouvel employeur est avant tout conçue pour protéger les salariés et empêcher que leur emploi ne disparaisse avec la perte du marché par l'entreprise sortante. Organiser le transfert des salariés permet d'assurer la continuité du service. Il s'agit, en l'espèce, de garantir la continuité du service de transport ferroviaire et de permettre aux nouveaux entrants

Nous avons, en commission, renforcé les droits des salariés de SNCF Mobilités qui seront transférés. Ces salariés bénéficieront du maintien des éléments essentiels du statut la garantie de l'emploi, l'affiliation au régime de retraite et un montant de rémunération équivalent, incluant l'ensemble des primes, indemnités, gratifications et allocations. Par ailleurs, nous avons souhaité favoriser au maximum le recours au volontariat des salariés, puisque pourront être volontaires pour rejoindre le nouvel entrant l'ensemble des salariés de la région concernée. Nous avons également prévu que, si le transfert implique un changement de région, les salariés pourront le refuser sans conséquence pour la poursuite de leur contrat de travail. Vous le voyez, mes chers collègues, cet article garantit aux salariés transférés un large socle de droits sociaux, loin, très loin des caricatures que nous pouvons parfois entendre. Ces caricatures font d'ailleurs mal au coeur parce que, franchement,

qui ont permis d'inscrire dans le texte à l'Assemblée nationale des principes forts en matière d'organisation des transferts de personnel en cas de perte de contrat par l'opérateur historique. Tout d'abord,

: garantie de l'emploi, régime spécial de retraite, garantie de rémunération, facilités de circulation, médecine de soins, logement. avons même été au-delà, dans le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, en organisant une véritable portabilité des droits, qui permet donc aux cheminots d'effectuer des mobilités volontaires en conservant ces mêmes garanties. Après l'adoption du texte à l'Assemblée nationale, j'ai souhaité poursuivre les concertations avec les deux organisations syndicales qui, sans être

Le scrutin est ouvert.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

Même si celle-ci est renouvelable, il n'y a aucune raison à notre sens de fixer un délai excessif pour les salariés de la SNCF qui seraient embauchés quelques mois avant le changement d'attributaire d'un contrat de service public pour que leur contrat soit transféré dans des conditions décentes. Quel est l'avis de

également compte de cette exigence. En ce qui concerne l'organisation collective du travail, il y aura un cadre au niveau de la branche, qui sera décliné au sein de chacune des entreprises.

un élément du réseau ferroviaire. Nous estimons, par principe, que ces structures doivent continuer à relever de Gares et Connexions, sous la responsabilité du groupe public ferroviaire intégré, et donc ne pas Nous sommes, par conséquent, opposés au recours au modèle « transporteur-intégrateur », qui permettrait de confier la gestion des gares au seul opérateur de ces infrastructures, et ce pour plusieurs raisons.

Nous estimons même que la démarche de contractualisation est contradictoire avec la volonté affichée d'unifier la gestion et l'exploitation des gares sous la responsabilité de SNCF Réseau, reconnaissance implicite du caractère déterminant d'infrastructure ferroviaire

ce qui implique d'intensifier encore une décentralisation qui s'opère déjà aujourd'hui, mais, hélas ! sans les ressources adéquates. Enfin, ouvrir la possibilité de confier l'exploitation des gares à un opérateur privé, même sous contrat avec une région, ne nous semble pas pertinent. Une gare, élément du réseau et partie intégrante du domaine public, ne peut être confiée à un opérateur privé. Nous proposons donc la suppression de cette possibilité d'intégration de la gestion des gares dans les contrats de service public. Quel est l'avis de la commission ? M. Gay a sa logique.

concerne également des salariés de l'opérateur sortant qui effectuent des prestations en gare. Actuellement, dans de nombreuses gares dites « monotransporteur où ne circulent que des trains gérés par SNCF Mobilités, la plupart des prestations en gare, comme l'accueil et l'information des voyageurs, sont assurées directement par SNCF Mobilités, et non par Gares et Connexions. Il serait, en effet, contre-productif que des agents de Gares et Connexions soient affectés dans ces gares où peu de trains circulent et où, par conséquent, l'accueil des voyageurs peut être assuré directement par l'opérateur de transport.

Il s'inscrit dans la volonté du Gouvernement d'instituer un cadre social de haut niveau applicable à l'ensemble des salariés. Il s'agit de s'assurer que les salariés transférés continueront de relever de la convention collective ferroviaire et bénéficieront de l'ensemble des stipulations qui seront négociées au titre de la construction d'un cadre social de haut niveau pour la branche. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à préciser que les contrats de travail des salariés transférés à un nouvel opérateur

certaines modalités à un décret et d'autres à la négociation de branche. Nous souhaitons que les organisations syndicales négocient sur l'ensemble des modalités de transfert, afin de garantir aux salariés transférés le maintien des droits sociaux acquis. Tous

Il ne vous aura pas échappé, cher collègue, que les partenaires sociaux ont déjà beaucoup d'autres sujets de négociation pour les mois à venir. Il va falloir accélérer ! Cet amendement vise à confier à un accord de branche, et non à un décret en Conseil d'État,

Gouvernement ? Il s'agit de définir le nombre de salariés affectés directement ou indirectement au service dans le cadre de l'organisation existante.

La notion de « maintenance lourde » n'a pas de définition précise et peut donc prêter à confusion. Plus généralement, il convient d'éviter de complexifier à l'excès le système ferroviaire par une ouverture partielle à la concurrence des prestations de maintenance du matériel roulant. Il convient, en particulier, d'exclure des solutions sous-optimales dans lesquelles l'activité de maintenance serait ouverte à la concurrence, alors même que les lots portant sur le transport de voyageurs n'atteindraient pas une dimension critique justifiant le transfert éventuel d'un centre de maintenance du matériel. Cette activité sera, par ailleurs, sujette à des creux de charge jusqu'en 2025. Elle doit donc faire l'objet d'un traitement particulier, visant à la maintenir intégralement au sein du groupe public ferroviaire, sous la forme d'un monopole régulé, accessible à l'ensemble des opérateurs. Pour illustrer mon propos,

imbriquées dans les services courants du transport régional.

et qu'il n'aura donc aucune conséquence sur le maintien du contrat de travail. Il appartiendra à SNCF Mobilités de formuler des propositions raisonnables permettant la poursuite de la relation contractuelle au sein du groupe public.

En effet, ce volontariat pourra concerner non seulement l'ensemble des salariés affectés, même très partiellement, au service transféré, mais également l'ensemble des salariés de la région affectés à d'autres services. Nous avons donc Nous avons donc fortement étendu le nombre de personnes pouvant se porter volontaires pour un transfert. Par ailleurs, le dispositif que nous avons inséré prévoit que les salariés qui ne sont pas affectés majoritairement au service transféré pourront refuser le transfert. Ils se verront dans ce cas proposer une offre de reclassement en priorité dans la région où ils habitent, et à défaut sur le reste du territoire national. si le nombre de volontaires est insuffisant, il est nécessaire d'avoir un mécanisme contraignant pour faire en sorte que le nouvel opérateur puisse disposer d'un nombre suffisant de salariés déjà formés pour exploiter le service ferroviaire.

à l'Assemblée nationale après concertations avec les organisations syndicales. Le Gouvernement était favorable à l'élargissement du périmètre du volontariat. Finalement, ne seraient concernés par un transfert obligatoire que les salariés les salariés majoritairement affectés au service et pour lesquels ce transfert ne supposerait pas de changement de résidence.

les cheminots et cheminotes sont évidemment attachés au service public, ils sont aussi profondément attachés à l'entreprise SNCF.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

La branche a besoin d'un socle social solide, qui assure son attractivité pour les salariés, sachant qu'une part importante des métiers du transport ferroviaire présentent des contraintes fortes pour les salariés. C'est une condition du développement d'un transport ferroviaire de qualité et sûr. Afin d'éviter le développement de pratiques de social allant à l'encontre des objectifs du présent projet de loi, il est nécessaire que les décisions qui seront prises dans le cadre de la convention collective prévalent sur d'éventuels accords d'entreprise portant sur les mêmes sujets. Une telle approche est cohérente avec le fait que, à défaut d'aboutissement de la négociation de branche, la législation prévoit que l'État intervienne par décret. Nous utilisons là une spécificité de la convention collective nationale de la branche ferroviaire, qui figure à l'article L. 1321-3-1

Dans le cas d'un refus de transfert d'un salarié dont le taux moyen d'affectation au service transféré sur les douze mois est inférieur à 50 %, l'article 2 prévoit actuellement que ce salarié se voie proposer une offre d'emploi dans la même région ou, à défaut, sur le territoire national de l'entreprise. Il nous paraît préférable de proposer une offre d'emploi alternative dans le département de résidence du salarié ou les départements limitrophes, car le dispositif actuel fait peser un trop grand risque de bouleversement de la vie du salarié et de sa famille. Cet amendement vise donc à mieux protéger les intérêts des salariés, tout en restant dans le cadre de la réforme.

continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui se substitue à elle, et ce pendant une durée d'un an. De plus, en l'absence de convention, il existe un socle de garanties, lequel porte exclusivement sur le niveau des rémunérations- ce dernier ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Avec cet

conservent les droits individuels résultant des conventions, décisions unilatérales, usages ou accords qui leur étaient applicables avant leur transfert au sein du nouvel opérateur. Cette disposition complémentaire doit inciter les partenaires sociaux à une contractualisation positive de substitution en cas de transfert d'activité. La survivance, au-delà de la durée légale d'un an, des droits individuels issus des accords, décisions et usages préexistants est sécurisante pour les salariés transférés. De plus, elle rend indispensable l'inventaire des droits et pratiques existants dans le périmètre de chaque lot transféré, afin de déterminer le cadre social nouveau qui devrait s'y substituer en tenant compte des enjeux économiques et sociaux propres au marché concerné. Cette mesure est nécessaire pour garantir la confiance et l'engagement des salariés dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, alors même

nous sommes face à une question d'équilibre. En vertu de cet amendement, quand, au sein du nouvel opérateur, un accord d'entreprise n'a pas été conclu, les droits individuels résultant des accords collectifs, des décisions unilatérales ou des usages en vigueur au sein de l'opérateur sortant seraient applicables aux salariés transférés. mesure reviendrait à transférer l'ensemble des droits individuels prévus par le statut et figurant dans les actes réglementaires et non réglementaires propres à la SNCF. Je songe, par exemple, aux usages locaux conférant des avantages aux salariés, lesquels sont nombreux et parfois non écrits. le rappelle, le texte issu des travaux de la commission garantit aux salariés de SNCF Mobilités l'essentiel des droits prévus par le statut : la garantie de l'emploi, l'affiliation au régime spécial de retraites et le maintien d'une rémunération identique comprise dans un sens large- englobe en effet la rémunération fixe, les primes, les indemnités, les allocations et les gratifications. Ces droits auront d'ailleurs vocation à être complétés par un accord de branche. En outre, chaque opérateur

le rappelle, ce projet de loi garantit aux salariés qui sont transférés un montant de rémunération, mais il n'oblige pas les nouveaux entrants à verser eux-mêmes de telles allocations aux salariés transférés.

tient notamment au fait que, compte tenu de la garantie de l'emploi dont bénéficient les salariés sous statut, la SNCF dispose de son propre régime d'assurance chômage, lequel est moins coûteux.

défavorable. L'amendement n° 135, quant à lui, vise à assurer le maintien du régime social et fiscal des allocations. Je comprends le souci d'assurer un traitement équitable des entreprises de la branche ferroviaire.

Il s'agit là d'un élément important de sécurisation dans les parcours personnels ; à charge des conventions collectives d'être suffisamment attractives pour que les salariés ne soient pas tentés de revenir au statut. Ce n'est pas aux salariés de la SNCF de payer les conséquences de la libéralisation. Il convient donc de garantir, pour celles et ceux qui ont d'ores et déjà été embauchés au statut, un véritable droit à réintégration, comme corollaire de la garantie de l'emploi. C'est tout le sens de notre amendement.

tout en veillant à l'équilibre entre leurs aspirations et les contraintes liées à l'exploitation du service public. Je me félicite de ce nouveau témoignage du dialogue fécond entre votre assemblée, le Gouvernement et les organisations syndicales, et j'ai le sentiment que les garanties apportées aux salariés en cas de transfert

En effet, le cas de défaillance du nouvel employeur, qui devra cesser son activité et licencier son personnel, est prévu dans le texte depuis l'adoption d'un amendement en commission tendant à faire supporter la charge aux autorités organisatrices, qui n'en ont pourtant pas les capacités.

l'avis de la commission

nous proposons que, en cas de changement d'employeur à l'initiative des salariés ou lors d'un transfert lié à un changement d'attributaire d'un contrat de service public, l'ancienneté de service acquise par les salariés dans les entreprises de la branche ferroviaire soit intégralement prise en compte pour l'appréciation des droits conventionnels et réglementaires en vigueur, dès lors que leur contrat de travail continue à être régi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. L'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire implique une mobilité accrue des salariés et de plus fréquents changements d'employeur au sein de la branche. Afin de favoriser cette mobilité, il apparaît nécessaire d'assurer aux salariés la prise en compte de leur ancienneté dans la branche, garante de leur expérience et de leur savoir-faire dans les métiers du ferroviaire. Le développement de parcours professionnels sécurisés dans la branche répond aux besoins des entreprises du secteur d'une fluidité de l'emploi, et facilite notamment leur capacité opérationnelle à assurer rapidement la prise en charge d'un nouveau service. La pleine reconnaissance de l'expérience du personnel recruté est essentielle. Elle doit aller de pair avec le développement des parcours de formation dans la branche. Tel est le sens de notre amendement. Quel est l'avis de la ? Cet amendement vise à prévoir que l'ancienneté de service acquise par les salariés soit prise en compte en cas de changement d'employeur. Il s'agit bien sûr d'une question importante, relative aux conditions de déroulement des carrières et d'évolution professionnelle au sein de la branche ferroviaire.

vous enverriez un message de confiance et de respect à toutes les personnes investies dans les négociations, qui planchent actuellement sur l'élaboration de la convention collective de la branche ferroviaire.

c'était un souhait très fort du président du Sénat, qui a eu des contacts importants avec les syndicats. Nous en avons eu également, avec le souci de les entendre et dans la limite, évidemment, de ce qu'il était possible de faire. On peut toujours considérer que ce n'est pas suffisant, mais

nous ne sommes pas pleinement satisfaits. En effet, notre position phare, la fin du recrutement au statut conditionnée à la négociation d'une convention collective ferroviaire nationale,

dans le prolongement des travaux de l'Assemblée nationale. Dès le départ, j'ai dit que, l'ouverture à la concurrence, je la souhaitais protectrice pour les cheminots. À partir des deux mois de concertation que j'avais engagés au début du mois de mars avec les organisations syndicales, nous avions pu inscrire des garanties importantes dans le texte voté par l'Assemblée nationale : la priorité donnée au volontariat, des garanties de haut niveau en cas de transfert, la garantie de l'emploi, le régime de retraite, la rémunération. Nous avions également introduit la portabilité des droits en cas de mobilité choisie au sein de la branche. Le Gouvernement a souhaité poursuivre les concertations. Deux organisations syndicales, qui ne partagent pas forcément les principes de la réforme,

le maintien de l'intégralité de la rémunération, l'élargissement du volontariat et la possibilité d'opter pour un retour au statut, à la SNCF.

Nous parlons donc déjà d'un service public sinistré. Pourtant, l'État, en faisant le choix de conventionner ces services dès 2010 et d'en devenir l'autorité organisatrice en 2011, avait envoyé un fort signal sur l'intérêt de ces lignes pour l'aménagement du territoire. tout en respectant totalement le règlement OSP, sur le fondement duquel l'exploitation des lignes d'équilibre du territoire a pu être qualifiée d' « obligation de service public susceptible de faire l'objet d'une compensation par l'État

L'aménagement du territoire et l'intérêt général qu'il recouvre répondent selon nous à une telle caractéristique spécifique. Ainsi, au lieu de privilégier l'ouverture à la concurrence, l'État pourrait choisir la voie de l'effort public pour ces lignes, en renforçant la convention avec SNCF Mobilités, l'opérateur historique du service public. Le développement de ces lignes passe non pas par un changement d'opérateur, mais par des investissements en termes de matériels roulants- l'État s'y est engagé -, d'infrastructures et de renforcement de l'offre. de l'offre. Or la contribution de l'État est prévue en baisse constante sur la période 2016-2020 ... Selon les modalités fixées par cet article, l'État pourra, entre 2019 et 2023, choisir la concurrence ou la poursuite des contrats avec la SNCF. À partir de 2023, l'obligation de mise en concurrence s'imposera à lui à l'issue de la dernière convention, dont la durée ne peut dépasser dix ans. La dernière convention signée entre l'État et SNCF Mobilités date du 17 février 2017

que leur exploitation par des opérateurs privés sera plus efficace et, surtout, maintenue, compte tenu de leur fréquentation souvent peu rentable ? Oui ! Ce service public a été décimé ces dernières années, je le répète, par une gestion purement comptable ayant conduit à des suppressions de ligne, notamment dans le service de nuit, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'intérêt social et environnemental de ces lignes. Pourtant, parlons clair : toute ligne supprimée a entraîné un report sur des bus ou sur la voiture individuelle. À l'heure de la COP24, c'est une aberration, tant on sait que le secteur des transports porte une lourde responsabilité dans l'émission de gaz à effet de serre ! Je réitère très solennellement notre opposition totale à cette vision à courte vue. Certes, il y a eu des engagements sur le renouvellement du matériel ferroviaire, mais cela n'est pas suffisant. Il faut changer de prisme et conventionner de nouvelles lignes, pour mieux répondre au défi climatique et aux besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens. La libéralisation du secteur entérine un changement de vision : le transport ferré est considéré non plus comme un outil de puissance publique, mais comme un secteur économique offrant un service avant tout marchand

Vous m'interrogez sur les intentions de l'État en tant qu'autorité organisatrice des services d'intérêt national. Celui-ci fera comme les régions, en tant qu'autorité organisatrice : si la qualité de service est au rendez-vous, l'État

soient ouverts à la concurrence, non pas en 2023, mais en 2033, afin de laisser à l'opérateur aujourd'hui en situation de monopole le temps de se préparer à cette évolution défavorable. Je vous rappelle les craintes, formulées par l'ARAFER, d'une multiplication des acteurs dans le secteur. L'effort de financement du réseau n'est

2023 en vertu du quatrième paquet ferroviaire, ne puisse pas être anticipée par l'État, comme le prévoit le présent article. Madame la ministre, vous pouvez au moins vous engager

Il ne faudrait pas laisser croire que des exceptions, qui auraient été négociées sous le précédent quinquennat, permettraient de satisfaire votre demande. Au demeurant, vous l'avez souligné, la date de renouvellement de ces contrats ou, en tout cas, la fin du contrat actuel, est fixée à 2020. Je le comme toutes les autres autorités organisatrices, l'État en tant qu'autorité organisatrice des services d'intérêt national n'a aucune raison de ne pas renouveler son contrat avec SNCF Mobilités, dès lors que la qualité de service est au rendez-vous. La rédaction actuelle du texte permet

en accord avec la présidente de région et présidente du STIF. Je le redis, personne n'envisage d'abandonner les trains d'équilibre du territoire. On est en train d'investir 3,7 milliards d'euros

je pense que l'on peut faire confiance à la SNCF pour offrir un service de grande qualité. Si ce service est à la hauteur des attentes des voyageurs, l'État n'aura évidemment aucune raison de ne pas renouveler la convention TET avec la SNCF

La question est simple : doit-on, oui ou non, prévoir des ressources nouvelles pour les régions, afin qu'elles développent leurs services ferroviaires, notamment dans le cadre de leurs nouvelles compétences, puisqu'elles récupèrent des anciennes lignes et, bientôt, des lignes à faible trafic ?

manquent de ressources pour organiser les mobilités de la vie quotidienne dans des territoires qui ne sont parfois pas desservis par le train,

comme les TER et les TET, le taux dévolu aux produits de première nécessité, soit 5,5 %, en considération de leur rôle social essentiel et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition énergétique.

Cette ouverture se fera à la découpe, contrat de service public par contrat de service public. Une telle démarche pose question au regard de l'unité du réseau et de la cohérence globale de son exploitation. vous nous dites que les régions sont majoritairement favorables à cette réforme. Aujourd'hui, oui, peut-être, mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas Ainsi, dans un avis de 2011, l'ARF estimait que les multiples réformes menées depuis 1997, afin de rendre la libéralisation possible, une désintégration du système, une multiplication des acteurs et une dilution des responsabilités, qui rendent l'ensemble incompréhensible. Multiplier les opérateurs sur un réseau en mauvais état et dont la gouvernance est en pleine crise, ne pourrait que créer des difficultés supplémentaires, voire porter atteinte à la sécurité des circulations. À nos yeux, cette analyse reste juste aujourd'hui. Les problématiques réelles qu'ont soulevées les autorités organisatrices portaient sur la vétusté des réseaux, le niveau des péages payés à SNCF Réseau et l'opacité de la SNCF. La libéralisation ne répond à aucun de ces enjeux de transparence et de financement du réseau ferroviaire. Au fond, cette ouverture à la concurrence n'a qu'un seul objectif : limiter le nombre de dessertes en faisant supporter le poids de cette décision Les régions, qui sont asphyxiées financièrement par les charges non compensées et la reprise d'un certain nombre de lignes, voient dans cet abandon une solution à une équation insoluble. L'État profiterait également de cette décision, puisque les dépenses de transport au titre des contrats de plan État-région diminueraient aussi. Il s'agit donc d'un jeu de dupes contre le service public ferroviaire et les usagers des transports. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

nous ne nous soyons pas encore compris sur le fait que les régions qui demandent cette ouverture à la concurrence ne le font évidemment pas pour réduire les dessertes. Cette ouverture à la concurrence se fait dans le cadre de contrats de service public. Je suis pour ma part certaine que les régions qui demandent cette ouverture à la concurrence le font pour obtenir un meilleur service, au meilleur coût, donc pour avoir encore plus de transports ferroviaires. Le Gouvernement

qui, pour le futur groupe public SNCF, va bien plus loin que les mesures prévues par la directive. En l'état, la rédaction de l'article empêcherait que le président de SNCF Réseau exerce également des responsabilités de dirigeant à la tête du groupe. à ce stade, nous ne souhaitons pas préjuger du choix de la future gouvernance du groupe. C'est la raison pour laquelle je vous propose une synthèse entre la stricte transposition de la directive et votre souhait d'une clarification des responsabilités au sein du groupe. Cet amendement tend ainsi à prévoir une incompatibilité entre, d'une part, toute responsabilité exercée dans la gestion du réseau ou des gares, et, d'autre part, toute responsabilité dans l'activité de transport ferroviaire. Pour le reste, la transposition du quatrième paquet ferroviaire, prévue par l'article 2 du projet de loi, permettra d'introduire, dans le droit national, les autres mesures de sauvegarde prévues par les textes européens. Quel est l'avis de

Or cet amendement tend à revenir sur la modification que nous avons opérée en commission pour conforter l'indépendance de SNCF Réseau. Dans le cadre d'une entreprise verticalement intégrée, comme le sera le groupe public unifié, avec une de tête et deux filiales, il convient de tout mettre en oeuvre pour s'assurer de l'indépendance du gestionnaire d'infrastructures, SNCF Réseau, vis-à-vis de l'opérateur de transports SNCF Mobilités. Il s'agit d'un enjeu important

Il ne faudrait pas, en effet, que la de tête puisse, à travers, par exemple, sa maîtrise de la politique des ressources humaines ou des services juridiques de groupe, influencer l'activité de SNCF Réseau pour servir les intérêts de SNCF Mobilités. Dans un tel cas, il n'y aurait plus de concurrence. il n'y aurait plus de concurrence. La question de la gouvernance est également cruciale. C'est pourquoi nous avons prévu, comme le recommande d'ailleurs le président de l'ARAFER, que nous avons entendu la semaine dernière, que les fonctions de membre de conseil d'administration ou de dirigeant de SNCF Réseau soient incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de dirigeant de la SNCF. Il serait effectivement inconcevable que, à l'avenir, dans le contexte d'ouverture à la concurrence, le président de SNCF Réseau puisse être également un dirigeant de la SNCF, comme c'est le cas aujourd'hui. Tel est le sens de l'amendement que nous avons adopté en commission, visant à renforcer le régime d'incompatibilité prévu à l'article 8 . Par conséquent,

Ces articles visent à organiser un transfert clefs en main aux régions des ateliers de maintenance et du matériel roulant. Nous sommes opposés à ce transfert, certes volontaire de la part des régions, mais qui contribue à dépecer et à vendre à la découpe l'entreprise historique.

le montant des investissements réalisés pour acquérir une flotte de matériel roulant ferroviaire constitue une importante barrière à l'entrée de concurrents. Transférer les matériels roulants et les ateliers de maintenance est donc l'une des conditions pour attirer de nouveaux opérateurs. C'est le seul intérêt de cette mesure.

comment faire le tri entre ce qui est transférable et ce qui ne l'est pas ? Il convient également de s'interroger sur l'avenir des politiques de maintenance, des processus industriels et de l'ingénierie ferroviaire gérés nationalement par les services de la SNCF, qui ont toujours démontré leur pertinence technique et leur capacité à assurer la sécurité et la qualité du matériel roulant. Au-delà de la perte de l'efficacité qualitative et économique d'une maintenance unifiée et pilotée de matière centralisée, comment pouvons-nous être assurés que, demain, cette maintenance morcelée, éclatée, ne se transformera pas en maintenance à plusieurs vitesses, mettant en péril la sécurité des usagers ? De nombreux points sont également à clarifier, notamment sur les conditions de transfert des personnels, la valeur des actifs ou la façon dont le coût de démantèlement des matériels roulants anciens sera pris en charge. En effet, les régions n'ont pas à supporter les conséquences financières de décisions prises antérieurement à la régionalisation du transport ferroviaire. Parce que cette reprise par les régions des matériels de la SNCF participera à l'affaiblissement de l'opérateur historique, nous proposons donc la suppression de cet article.

J'entends bien que nous ne sommes pas d'accord sur l'objectif d'ouverture à la concurrence, mais les nouveaux opérateurs, tout comme la SNCF,

Dans la rédaction actuelle, seules les autorités organisatrices communes, les régions, sont tenues de le faire, alors qu'elles subissent déjà de plein fouet la baisse des dotations de l'État et qu'elles devront faire face à une réorganisation importante

précision figure à l'alinéa 3 de l'article 2 : « L'autorité organisatrice prend en charge les coûts de démantèlement des matériels roulants qu'elle ne reprend pas à proportion de la durée d'utilisation de ces matériels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, déduction faite des provisions qui lui auraient été déjà facturées ». Cela me paraît clair ! C'est du

Merci,